également à remercier le Premier ministre, actuellement en déplacement en Chine, vous-même, monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, et l'ensemble des ministres, ainsi que les membres des cabinets ministériels, en particulier les conseillers parlementaires, grâce auxquels le dialogue républicain entre l'exécutif et la Haute Assemblée a pu se nouer de manière positive et fructueuse. Les travaux en séance plénière seront suspendus à l'issue de l'après-midi. Pour autant, Pour autant, le Sénat continuera à travailler au sein des groupes, des commissions permanentes, des délégations, des commissions d'enquête, des missions d'information, des groupes de travail ou d'études,

les droits des victimes, me conduisent à vous interroger, encore une fois, sur l'action du Gouvernement en matière de lutte contre la pollution de l'air, cette dernière demeurant la première préoccupation environnementale et sanitaire des Français. Alors que la France est de nouveau sous la menace de poursuites judiciaires devant les instances européennes pour son inaction dans ce domaine, alors que le rapport de la commission d'enquête du Sénat a estimé,, le coût annuel de la pollution de l'air à 101,3 milliards d'euros, il m'apparaît essentiel d'évoquer la souffrance humaine,

Devant ce fléau et le vide juridique qui l'entoure, il est grand temps que l'État prenne enfin ses responsabilités. En effet, force est de constater que rien n'est fait, aujourd'hui, pour venir en aide aux victimes. Madame la ministre, cette injustice sanitaire est souvent aussi une injustice sociale. Ma question est simple : à défaut de sanctionner les pollueurs, l'État va-t-il enfin reconnaître et prendre en charge les victimes de la pollution de l'air en France ?, par ailleurs, du secrétariat général à l'aide aux victimes créé la semaine dernière ? Excellente

d'État chargé de l'industrie. Arc International est le premier groupe verrier du monde. C'est aussi la plus grosse entreprise industrielle du Pas-de-Calais, qui emploie encore plus de 5 000 salariés. a failli disparaître en décembre 2015. Il a fallu une intervention forte de l'État et beaucoup de courage aux salariés pour permettre sa reprise par le groupe américain PHP. Les banques françaises ont dû effacer l'essentiel du passif et l'établissement public foncier a amené des liquidités à l'entreprise. L'exercice 2016 a redonné espoir aux salariés : finis les plans de départs volontaires, la menace de licenciements massifs ! L'entreprise s'est réorganisée, elle a retrouvé son dynamisme. Elle s'est d'ailleurs lancée dans une politique d'investissements massifs, financés par le recours à un consortium alliant un fonds souverain russe et la Caisse des dépôts et consignations, qui

Mais, depuis, rien ne semble se passer comme prévu. Aujourd'hui, l'entreprise est dans une mauvaise passe. Le fonds souverain russe semble réticent à débloquer la deuxième tranche de 50 millions d'euros, le propriétaire américain ne semble pas décidé à remettre la main à la poche, et c'est l'avenir du groupe qui est de nouveau menacé. Comment en est-on venu à livrer les destinées d'un fleuron de l'industrie française à un fonds d'investissement américain, puis à un fonds souverain russe ?

pour assurer la pérennité et le développement d'Arc International ? Quel rôle le Comité interministériel de restructuration industrielle peut-il jouer pour aider le groupe à obtenir l'appui de la Banque européenne d'investissement ? Il y a urgence, monsieur le secrétaire d'État, à répondre à ces questions

et nous avons été informés, la semaine dernière, de la nomination d'un nouveau directeur général d'Arc France, M. Tristan Borne, qui devrait prendre ses fonctions le 3 avril prochain.

certains réseaux sociaux ont été manipulés la technique des, ces fausses informations qui circulent sur la Toile et sont relayées indéfiniment par des internautes virtuels.

Monsieur le ministre, pourriez-vous nous rassurer, ou mieux encore nous garantir que tout sera mis en oeuvre pour que les prochaines échéances électorales se déroulent dans les meilleures conditions de transparence et de régularité ?

Depuis maintenant seize ans, l'ANDRA exploite un laboratoire souterrain, implanté en Meuse et en Haute-Marne, à 490 mètres de profondeur. Les recherches démontrent la faisabilité du projet. En 2006, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après un débat public, le Parlement a entériné le choix du stockage en couche géologique profonde. En 2013, un deuxième débat public a eu lieu. Ses conclusions ont alimenté les dispositions de la loi du 25 juillet 2016 relatives aux modalités de création de CIGEO et à la réversibilité. En janvier 2016, la ministre de l'environnement a arrêté le coût objectif du projet à 25 milliards d'euros. Par ailleurs, le stockage en couche géologique profonde constitue une référence internationale scientifiquement reconnue au bénéfice de l'industrie française. Un projet aussi complexe peut toutefois légitimement susciter des interrogations et des inquiétudes. Des Des oppositions démocratiques s'expriment et enrichissent le débat. Cependant, l'ANDRA se voit confrontée depuis plusieurs mois à des manifestants d'une agressivité de plus en plus radicale. radicale. Ils usent de moyens illégaux en occupant des propriétés privées et en dégradant des installations publiques. Le week-end dernier, des affrontements extrêmement violents ont eu lieu, marqués par des jets de pierres sur les forces de l'ordre. Je voudrais d'ailleurs souligner la maîtrise de la situation par la gendarmerie, sous la responsabilité de Mme la préfète de la Meuse. Monsieur le ministre, il me semble indispensable que vous confirmiez le soutien de l'État, nécessaire au déroulement normal de ce projet, et que vous rassuriez les populations locales, qui subissent les troubles suscités par ces casseurs, en prenant toutes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre et en déférant devant la justice les auteurs de ces troubles.

à la mouvance écologiste radicale contestent ce projet par la violence et souhaitent installer sur place ce qu'ils appellent une « zone à défendre à défendre », ou ZAD. L'État a engagé une procédure judiciaire visant l'occupation illégale du site. La violence des opposants, vous avez eu raison de le rappeler, s'est particulièrement manifestée la semaine dernière. En effet, du mardi 14 au dimanche 19 février 2017, la mouvance antinucléaire d'opposition au projet CIGEO a conduit une semaine d'action pour soutenir les occupants du bois Lejuc.

Ce quinquennat s'achève dans une situation internationale très préoccupante, à la fois complexe, confuse et dangereuse

seraient tombés aux mains des terroristes ou auraient connu des massacres de masse. C'est le Président de la République qui a assumé, au nom de la France, la responsabilité d'intervenir. À l'heure où les forces irakiennes mènent une offensive pour libérer la partie occidentale

la Syrie, la France a la conviction que seule une solution négociée, fondée sur une transition politique, édifiée sur la base du communiqué de Genève et de la résolution 2254 du Conseil de sécurité de ramener la paix. Après les résultats en demi-teinte des réunions d'Astana, les discussions ont repris aujourd'hui à Genève. À cet égard, nous apportons notre plein soutien aux efforts de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies, M. Staffan de Mistura. La France est également engagée au Proche-Orient pour tenter de relancer un processus politique. Dans le contexte actuel, l'initiative du ministre des affaires étrangères, qui a réuni plus de soixante-dix pays et organisations internationales à Paris, le 15 janvier, était non seulement utile, mais nécessaire, pour défendre la solution à deux États. Oui, nous sommes engagés en Méditerranée ! Oui, nous avons fait en sorte que l'Europe s'engage aux côtés de la Tunisie et qu'elle se mobilise pour aider à élaborer une solution à la crise libyenne ! Oui, nous avons respecté nos engagements concernant la loi de programmation militaire ! Nous les avons même rehaussés,

foncier et d'établissement rural, les SAFER, qui disposent des outils adéquats pour limiter le risque d'accaparement des terres agricoles par des sociétés étrangères, comme l'a si bien souligné mon collègue Alain Bertrand la semaine passée.

fragilisés, comme l'a souligné le député Pierre Aylagas dans une question écrite. Au déséquilibre économique subi s'ajoutent le pillage du potentiel de production, ainsi que des préjudices sanitaires et environnementaux.

la fin de la régulation des plantations viticoles dans l'Union européenne. Vingt ans après ... Nous l'avons sauvée au travers de la réforme de la PAC de 2013.

et une partie du nord des Pyrénées-Atlantiques. Sous quinze jours, tous les palmipèdes de ce périmètre seront abattus. Parallèlement, une interdiction de mouvements a été décidée pour l'ensemble des Landes et du nord des Pyrénées-Atlantiques. Il n'y a pas d'autre stratégie possible, la vaccination ne permettant pas de stopper la diffusion du virus. Les remises en place de palmipèdes ne seront possibles que d'ici à la fin du mois de mai, mais les gallinacés peuvent d'ores et déjà être remis en place dans les zones stables. les zones stables. Concernant l'indemnisation, là encore l'État sera au rendez-vous. Pour l'amont de la filière, les premiers versements interviendront en mars pour les éleveurs ayant subi un abattage et les pertes économiques dues aux restrictions de mouvements seront indemnisées au printemps.

Les mesures devront bien sûr être adaptées aux différents types de production et aux capacités d'investissement des acteurs, notamment des éleveurs. En tout état de cause, monsieur le sénateur, nous veillerons à préserver la diversité des situations et des modèles.

les 300 000 Français établis au Royaume-Uni, et au-delà les 3 millions d'Européens vivant outre-Manche, n'ont reçu aucune assurance sur leur statut de la part des autorités britanniques. La situation devient de plus en plus anxiogène, sur fond de xénophobie ambiante et décomplexée, nourrie par les atermoiements de Theresa May, qui ne veut pas déplaire à des tabloïds qui font de la haine de l'Europe leur fonds de commerce. Les Européens ne se sentent plus bienvenus.

Les employeurs refusent désormais de prendre le risque d'embaucher en CDI des ressortissants de l'Union européenne. Ceux-ci vivent cette discrimination avec beaucoup d'amertume. Lundi dernier, avec Patricia Connell et Nicolas Hatton, nos élus consulaires du Royaume-Uni, j'étais aux côtés de milliers de manifestants devant Westminster à l'appel du mouvement The 3 Million, qui exige une clarification, dès à présent, du statut des 3 millions de citoyens de l'Union européenne résidant au Royaume-Uni. Ces derniers refusent de servir de monnaie d'échange lors des futures transactions. Vendredi dernier, le Premier ministre a rencontré Theresa May. Qu'avez-vous fait pour que les droits des Européens établis au Royaume-Uni soient préservés ?

Nous pourrions leur accorder, immédiatement et sans contrepartie, le maintien de leur statut de citoyen européen jusqu'à la fin de leur vie. Ainsi, le Brexit n'aurait pas d'effet sur eux. Une telle démarche placerait le Gouvernement britannique devant ses responsabilités. Il ne pourrait plus se servir des Européens installés au Royaume-Uni comme d'une monnaie d'échange lors de futures négociations.

Je voudrais partager l'état des lieux qu'est en train de dresser la commission des lois du Sénat, qui enquête depuis plus de six mois sur la situation de la justice française. Celle-ci est grave. J'évoquerai quelques indicateurs qui sont, hélas ! éloquents : le

la moitié seulement des condamnations reçoivent un commencement de mise à exécution dans l'année qui suit le prononcé. La politique pénale est un fiasco Vous avez renoncé à créer des places de prison et souhaitez vider les prisons en privilégiant une nouvelle politique, celle de la contrainte pénale. la contrainte pénale ne représente que 1 000 décisions par an. En revanche, nos magistrats veulent être sévères : ils ont prononcé 130 000 condamnations en 2016 ; n'est-ce pas là un désaveu cinglant ?

à une saturation de nos prisons, qui accueillent 68 000 détenus pour 58 000 places. N'est-il pas temps de dresser le constat d'échec de cette politique ?

Il y a un mois, à Saint-Herblain, le petit David, âgé de huit ans, est décédé après avoir subi des actes de torture et de barbarie commis par sa mère et son compagnon. Quelques jours plus tard, à Vitry-sur-Seine, le jeune Oumar, quinze a succombé aux coups de ceinturon infligés par son beau-père. Le 6 février dernier, à Aire-sur-la-Lys, le jeune Yannis, cinq ans, est mort après avoir été puni pour avoir fait pipi au lit, frappé par son beau-père qui l'a forcé à courir dans le froid en pleine nuit.

Devant ces drames, notre société ne peut rester aveugle et sourde. Cette violence, nous le savons, recouvre des réalités diverses : violences physiques, violences sexuelles, violences psychologiques. que ces sévices ne se terminent pas toujours par un décès, leurs conséquences sont graves pour les victimes. Le coût social du traitement médical et psychologique de ces jeunes et de ces adultes en devenir se chiffre en milliards d'euros.

de la liberté éducative, du rôle de l'école, des droits de l'enfant, de l'éducation à la sexualité et de la responsabilité dont chacun d'entre nous

Il faut conclure, madame la ministre. Il devient alors impossible, pour qui que ce soit, d'établir la différence entre la violence quotidienne, les punitions corporelles, le droit de correction et les maltraitances faites aux enfants. Je présenterai la semaine prochaine le premier plan de lutte interministériel contre les violences

Contrairement à vos annonces, le déficit de la sécurité sociale sera d'environ 4 milliards d'euros en 2017. La seule amélioration enregistrée est liée essentiellement à la réforme du régime des retraites réalisée par vos prédécesseurs, que vous aviez combattue. au regret de devoir constater que vos réformes successives de la santé ont été aussi dogmatiques que bureaucratiques. Le niveau de remboursement des patients a baissé avec les contrats dits « responsables ». Le malaise à l'hôpital n'a fait que croître, et en décourageant la médecine libérale, vous avez favorisé le développement des déserts médicaux. La baisse des allocations familiales a été un coup dur porté aux familles. Dans le même temps, vous n'avez pas su faire prendre au pays le virage du XXI siècle : nous en avons débattu ici

Le temps du bilan est venu. Ne pensez-vous pas que, face à la situation sociale inquiétante que connaissent les Français, face à la désespérance de beaucoup de nos compatriotes, il serait temps de faire résonner vos paroles avec la réalité ?

Durant la législature précédente, 280 000 emplois avaient disparu ! Et combien de chômeurs de plus ? Le nombre des demandeurs d'emploi a augmenté de 500 000 durant cette législature. C'est trop,

La séance est reprise. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat qu'il a été saisi le 23 février 2017, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante députés, de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Le texte de la saisine est disponible au bureau de la distribution. Acte est donné de cette

de loi. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la présente proposition de loi répond à une forte attente de nos territoires, dont les élus appréhendent le transfert des compétences « eau » et « assainissement Comme vous le savez, le régime d'attribution des compétences « eau » et « assainissement », dont l'exercice est complexe et hétérogène dans les territoires, a été sensiblement modifié par la loi NOTRe. Antérieurement à l'adoption de ce texte, l'assainissement figurait au rang des compétences optionnelles, un des sept groupes relevant du choix des communautés de communes. La compétence « eau », facultative, pouvait être librement transférée à l'intercommunalité par décision des communes membres, à la majorité des deux tiers. Dans un objectif de renforcement de l'intégration communautaire, la loi NOTRe a élargi le bloc des compétences obligatoires des communautés de communes. Celui-ci comprend désormais l'eau et l'assainissement, le transfert étant organisé en deux temps d'ici au 1 janvier 2020. aux termes du droit en vigueur, les services de l'eau et de l'assainissement seront obligatoirement pris en charge par les communautés de communes. Avant cette échéance, la loi NOTRe a prévu des mesures transitoires. Les communautés de communes existant à la date de publication de la loi auront jusqu'au 31 décembre 2017 pour se conformer aux nouvelles dispositions. Lors des débats sur la loi NOTRe au Sénat, Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, corapporteurs du texte, s'étaient opposés à la démarche du Gouvernement visant à créer de nouvelles compétences obligatoires pour les communautés de communes. L'amendement du Gouvernement prévoyant la création de ces nouvelles compétences obligatoires avait suscité une vive opposition transpartisane au Sénat. Notre assemblée avait donc adopté en deuxième lecture un texte dans lequel l'eau et l'assainissement avaient été classés au rang des compétences optionnelles des communautés de communes, afin de faciliter leur fonctionnement et au nom au nom du principe de subsidiarité. Aujourd'hui, le transfert de ces compétences suscite de nombreuses difficultés au sein de nos territoires, ce qui nous rappelle la nécessité, en matière de réformes territoriales, de faire preuve de pragmatisme.

exerçant la compétence « eau » en gestion directe- c'est-à-dire en régie -fournissent déjà l'eau à un coût relativement faible pour les usagers et la collectivité. Comme vous le savez, la gestion des services de l'eau et de l'assainissement est tributaire de nombreuses considérations géographiques, matérielles et techniques : il s'agit souvent d'exploiter un réseau physique La composition et l'organisation du réseau d'eau et d'assainissement dépendent nécessairement des spécificités, notamment physiques, des territoires. Or la loi n'est pas toujours en mesure d'anticiper les difficultés propres à de tels bouleversements dans l'exercice des compétences des communes. Sur nos territoires, communes et syndicats exercent actuellement les compétences « eau » et « assainissement » de manière efficace et économique, dans l'intérêt des citoyens et, surtout, en tenant compte des contraintes techniques et géographiques liées à cet exercice. Doit-on, Doit-on, au nom du seul renforcement de l'intercommunalité, mettre fin à ces pratiques adaptées à nos territoires ? si c'est dans la bonne direction ». Or la direction prise avec la loi NOTRe, sur cette question, n'est pas conforme à l'intérêt de nos concitoyens. Le texte dont nous allons débattre a pour objet de remédier aux difficultés créées par ce transfert de compétences. Il vise à limiter les effets des dispositions de la loi NOTRe relatives à l'eau et à l'assainissement en supprimant le caractère obligatoire, à compter du 1 janvier 2020,

cette proposition de loi permettra de conforter la commune comme cellule de base de la démocratie locale. Comme je l'ai indiqué précédemment, les spécificités des compétences « eau » et « assainissement » font de la commune l'échelon territorial le plus à même de les exercer avec efficacité. D'autre part, ce texte vise à remédier aux difficultés pratiques liées à ce transfert de compétences. Il procède d'une simple application du principe de subsidiarité, selon lequel une compétence doit être exercée par l'échelon le plus pertinent, en l'occurrence le plus proche des usagers.

de leurs compétences à l'intercommunalité. En application de ces principes, il doit revenir aux communes de choisir le niveau d'exercice des compétences « eau » et « assainissement ». Un transfert rationalisé de ces compétences implique que les communes soient libres d'en déterminer le rythme et le calendrier. Le maintien du caractère optionnel de ces compétences répond à un impératif de pragmatisme et de flexibilité pour les communes. Cela n'affecte pas les chantiers de transfert déjà en cours dans de nombreuses communautés de communes. Ce texte est d'autant plus nécessaire que, comme l'a souligné notre rapporteur, l'eau représente un enjeu de développement territorial. Il serait en effet peu opportun de retirer à des syndicats cette compétence au profit d'une intercommunalité n'ayant aucun savoir-faire en matière de gestion de l'eau et d'assainissement ne présentant parfois aucune cohérence en termes de périmètre.

de bénéficier de plus de temps et de plus de flexibilité dans l'exercice complexe de ces compétences, notamment en zone rurale ou de peuplement irrégulier. Le Sénat, en adoptant ce texte,

l'Association des maires de France observe que « l'organisation des services de l'eau répond à des logiques de qualité et de disponibilité de la ressource qui dépasse les frontières administratives ». La question

de coûts supplémentaires pour l'usager, mais également pour les budgets annexes de l'eau, qui sont souvent, dans les petites communes rurales, les seuls budgets excédentaires.

a en effet confié de nouvelles responsabilités aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération. Celles-ci sont compétentes, depuis le 1 janvier dernier, en matière de prévention et de gestion des déchets ménagers, de développement économique- je pense en particulier à l'ensemble des zones d'activité -ou encore d'accueil des gens du voyage. Au 1 janvier prochain, elles seront également chargées de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, au titre de la compétence GEMAPI. La loi NOTRe a enfin prévu, et c'est le coeur de notre sujet, le transfert à titre optionnel en 2018, puis obligatoire en 2020, des compétences « eau potable » et « assainissement » à l'ensemble des communautés de communes et des communautés d'agglomération. La proposition de loi discutée aujourd'hui vise à revenir sur ce transfert, qui resterait seulement optionnel. En revanche, le texte ne remet pas en cause les dispositions de la loi NOTRe concernant les communautés d'agglomération. Mesdames, messieurs les sénateurs, de quoi parlons-nous précisément ? Le service public d'eau potable se décline en deux types de missions : une mission obligatoire de distribution de l'eau potable aux usagers et des missions facultatives de production, de transport et de stockage. Le service public d'assainissement comporte, quant à lui, deux volets distincts : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif.

qui ont conduit le Gouvernement à proposer au Parlement de confier ces services publics de première nécessité à l'échelon intercommunal. Selon le dernier recensement réalisé par l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement, il existe environ 35 000 services d'eau et d'assainissement

dans près de 80 % des situations, la commune reste l'autorité organisatrice du service. Ces quelques chiffres témoignent de l'extrême atomisation de notre organisation locale. Transférer aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération ces compétences permettra donc de mutualiser les moyens techniques et financiers indispensables à un service public de qualité.

En outre, le transfert à l'intercommunalité permettra de disposer d'une assise financière accrue, dans un contexte global difficile pour les finances publiques, et alors que les services d'eau potable et d'assainissement connaissent ces dernières années un effet de ciseau, entre des ventes d'eau en diminution et des charges d'exploitation qui continuent d'augmenter. Par définition, les regroupements faciliteront une approche plus globale de la gestion de la ressource en eau, notamment de ses enjeux environnementaux. Cette gestion intercommunale doit ainsi constituer le trait d'union entre ce que l'on appelle communément le « petit cycle » et le « grand cycle » de l'eau, d'autant que

une mesure d'équité et de justice. Est-il normal que les tarifs et la qualité du service public de l'eau diffèrent autant d'un village à l'autre ? l'autre ? L'eau potable et l'assainissement constituent des services publics de première nécessité, comme l'électricité. Sur le même modèle, on pourrait même soutenir -certains ont eu le courage de le faire -la mise en place de tarifs nationaux. La réforme territoriale va assurer une cohérence à l'échelle intercommunale ; c'est déjà une avancée que l'on ne saurait combattre. Les transferts proposés vont conduire à de profondes évolutions, je ne le nie pas, sources parfois d'inquiétudes sur le terrain. Je reçois de nombreux courriers qui en attestent. Toutefois, le calendrier prévu permet de se préparer dans de bonnes conditions.

de ces compétences ne se traduira pas nécessairement du jour au lendemain par l'harmonisation du service et des tarifs. Bien évidemment, cela doit rester un objectif à atteindre dans des délais raisonnables. raisonnables. Les contrats en cours continueront à produire leurs effets jusqu'à leur échéance, sauf décision négociée par l'intercommunalité avec les tiers concernés. Par conséquent, et même si l'on peut le regretter, des tarifs différenciés pourront exister. Ce n'est pas exactement ce que l'on appelle un institutionnel, convenez-en. Je souhaiterais enfin dire quelques mots sur le devenir des syndicats intercommunaux existants. Un certain nombre d'entre eux ont certes vocation à disparaître. Mais, là encore, la loi répond un objectif de mutualisation des moyens, tout en tenant compte de la nouvelle carte intercommunale issue des travaux des commissions départementales de coopération intercommunale. Il ne s'agit pas de supprimer les outils existants permettant de répondre aux enjeux que je viens de préciser. Ainsi, comme le prévoit la loi NOTRe, dans les syndicats dont le périmètre recouvre tout ou partie du territoire de trois EPCI à fiscalité propre au minimum, les communautés de communes se substitueront automatiquement à leurs communes membres. Les grands syndicats techniques seront donc préservés. Je pense d'ailleurs que la constitution de grands syndicats départementaux peut représenter un modèle d'organisation pertinent. Certains

Il est regrettable de vouloir remettre en cause une disposition majeure de ce texte, particulièrement dans le calendrier proposé. Le 16 juillet 2015, en effet, le projet de loi était adopté par le

! Je m'étonne toujours de constater, plus d'un an après mon arrivée au ministère, la volonté de nombreux parlementaires de remettre en cause les dispositions fondamentales d'une loi votée

! Mesdames, messieurs les sénateurs, le transfert aux communautés de communes des compétences « eau potable » et « assainissement » est parfaitement cohérent. Il répond à un enjeu essentiel assurer un service public de qualité, sur le long terme, à l'ensemble de nos concitoyens, et aller vers davantage d'équité et de justice. Dans ces conditions, vous l'aurez compris, le Gouvernement ne peut être que défavorable à cette proposition de loi.

Madame le président, monsieur le ministre, chers collègues, la loi NOTRe et tous les autres textes qui l'ont précédée

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les collectivités ont besoin de stabilité pour mettre en oeuvre les politiques publiques dont elles ont la charge. Nous partageons ainsi la volonté affichée par les auteurs de cette proposition de loi de ne pas les contraindre inutilement en rendant obligatoires des transferts de compétences, en l'occurrence les compétences « eau » et « assainissement

Il est ainsi aujourd'hui de bon ton, pour le groupe Les Républicains, de se poser comme le défenseur des libertés locales. Certes, lors de l'examen de la loi NOTRe, le Sénat a fait bloc, toutes tendances politiques confondues, pour refuser le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement ». Pour autant, il faut tout de même rappeler que la logique de dévitalisation des communes et de leur asphyxie financière a été amorcée en 2010, lorsque l'actuel candidat à l'élection présidentielle François Fillon était Premier ministre. En effet, la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a ouvert la voie au territorial que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agissait, à l'époque, de prévoir le rattachement à une intercommunalité des dernières communes isolées, la suppression des syndicats intercommunaux prétendument obsolètes et la rationalisation du périmètre des EPCI. Pour ce faire, des pouvoirs importants étaient donnés aux préfets, au rebours de l'esprit même de la décentralisation. Ensuite, alors que ce quinquennat devait marquer une rupture, les lois MAPTAM et NOTRe sont venues amplifier ce mouvement de dévitalisation de l'échelon communal, en vue de parvenir à l'effacement et à la disparition des communes. Notre groupe est le seul groupe parlementaire à avoir conservé une position cohérente de défense des communes comme lieux vivants de la démocratie, en se prononçant pour des EPCI librement choisis, fondés sur des projets communs et partagés.

Par ailleurs, la proposition de loi prévoit un champ d'application bien réduit. Elle ne concerne que les communautés de communes, ignorant les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. Elle ne s'adresse ainsi qu'aux territoires ruraux, alors que la problématique est identique en milieu urbain. Le positionnement adopté aujourd'hui par le groupe Les Républicains indique clairement que nous sommes entrés en campagne pour les élections sénatoriales. Redonner du pouvoir aux collectivités locales exige en premier lieu de leur donner les moyens d'assumer leurs compétences dans de bonnes conditions. Or la baisse généralisée des dotations a rendu la tâche particulièrement ardue pour les communes. Pour notre part, nous proposons de mettre fin à cette asphyxie financière. Sur le fond, nous partageons la volonté affichée par les auteurs de cette proposition de loi.

Nous voyons en outre dans la marche forcée vers des intercommunalités de taille géante, absorbant l'ensemble des compétences communales, une démarche antidémocratique et contre-productive, puisqu'elle éloigne les lieux de pouvoir de nos concitoyens. Or le contrôle de la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement doit pouvoir être exercé par nos concitoyens, au plus proche des réalités. Nous voyons également dans ce transfert obligatoire un manque d'efficacité évident. Il faut laisser aux communes la souplesse de pouvoir s'associer librement au niveau du bassin hydrique, sans multiplier les transferts de compétences en cascade, qui, de plus, rendent totalement illisible l'action publique. Par ailleurs, nous craignons que ces regroupements engagent un accroissement des délégations de service public, alors même que nous observons un important mouvement en faveur d'un retour à une maîtrise publique des services de l'eau et de l'assainissement. Les régies publiques disposent d'un incontestable savoir-faire dans la défense de l'intérêt public et pour garantir aux usagers des prix accessibles pour tous, la plupart d'entre elles appliquant une tarification graduée. Tout bouleversement institutionnel autoritaire aiguisera les velléités du secteur privé de reprendre des marchés, avec les risques d'augmentation du prix de l'eau que cela induirait. Il ne s'agit pas d'un enjeu mineur, car le budget cumulé des syndicats de l'eau atteindrait près de 18 milliards d'euros. Ces transferts de compétences obligatoires rebattent donc les cartes au détriment de l'intérêt public et des usagers. Pour notre part, nous considérons qu'il convient de faire confiance aux élus locaux pour atteindre une plus grande efficacité dans la mise en oeuvre des politiques publiques dont ils ont la charge.

ne pas le voir. Que faut-il faire de la loi NOTRe et, accessoirement, de la loi MATPAM, au regard de leurs résultats sur le terrain, et plus encore peut-être de ceux à venir Certainement pas ! ... au risque d'ajouter encore à la confusion et de retarder un peu plus encore la remise en route administrative du pays, ce qui ne semble pas être la position dominante ? Faut-il, au contraire, continuer à composer, au risque de perpétuer ce tombeau bureaucratique de la démocratie locale ?

Ainsi, pour moi, il est impératif d'arrêter la prolifération des métropoles et le processus de leur transformation en communes dès lors que les conseillers métropolitains seront élus directement par la population. également impératif d'arrêter la vampirisation des départements par les métropoles, ce qui pose la question du mode d'exercice des compétences départementales par ces dernières : délégation ou transfert définitif ? Il est impératif aussi, si l'on entend redynamiser les communes rurales, les villes petites et moyennes, de redonner aux départements les moyens légaux et financiers d'assumer la « solidarité territoriale » dont ils ont déjà en principe la charge. Quant aux intercommunalités issues de la loi NOTRe, il faudrait au minimum continuer à prévoir des assouplissements en termes de compétences obligatoirement transférées et de représentation des communes. Il faudrait aussi, pour redonner sa place à la négociation locale, améliorer l'articulation entre communautés et syndicats, ce qui suppose que l'on renonce à l'objectif d'une réduction massive du nombre de ces syndicats. Enfin, s'agissant des intercommunalités « XXL », il paraît difficile d'échapper à une remise à plat de leur mode de constitution et de leur fonctionnement. On risquerait autrement de voir émerger des formes d'organisation n'ayant plus grand-chose à voir avec la démocratie. Je pense à ce qu'il restera de celle-ci avec des conseils pléthoriques et la délégation systématique des choix réels à des cénacles choisis, quand ce n'est pas à la bureaucratie communautaire S'agissant du présent texte, il est bien évident que le RDSE le votera, parce qu'il correspond à sa philosophie de l'intercommunalité, qui doit être essentiellement assise sur le volontariat, parce qu'il permettra de mieux coller au terrain. S'il existe des intercommunalités, communautés de communes et aussi communautés d'agglomération, dont la ressource en eau et son traitement dépendent obligatoirement d'actions coordonnées et de financements collectifs, il en est d'autres,

la gestion est souvent concédée. Pourquoi mettre à mal un mode de gestion qui donne satisfaction ? Parce que l'avenir est aux grandes organisations, nous susurrent les zélotes de la modernisation libérale Ils se trompent : l'avenir est à la coopération volontaire, seule capable de mobiliser initiatives et volontés, et de permettre l'émergence d'un idéal civique, cet idéal civique perdu dans le sable des modernisations

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier François Zocchetto d'avoir été, avec Bruno Retailleau, à l'origine de ce texte. On a le sentiment que la voix des communes a été entendue. Jusqu'à présent, les communes membres d'une communauté de communes pouvaient ou non choisir d'opérer ce transfert de compétences selon un critère totalement ignoré par les lois NOTRe et MAPTAM : le critère optionnel, le critère du choix, choix bien évidemment sous-tendu par l'intérêt général des habitants.

précitées. Bon sens, pragmatisme, arguments d'essence girondine battus en brèche par l'esprit aveugle et monolithique d'une rationalisation jacobine. Il y aurait beaucoup à dire, mais je ne dispose que de trois minutes Dans le cas qui nous occupe, celui des communautés de communes, les compétences « eau » et « assainissement » s'exercent le plus souvent au sein de zones rurales au peuplement irrégulier, où les communes ont organisé ces services à faible coût.

Ces communes, souvent peuplées d'agriculteurs dont nous connaissons les graves difficultés, sont pauvres pour la plupart d'entre elles. Les obliger à opérer ce transfert de compétences serait les contraindre de manière inacceptable. Les transferts autoritaires des compétences communales prévus par les lois NOTRe et MAPTAM n'ont tenu compte ni de l'existant ni de l'opinion des maires et des élus communaux. Pourquoi détruire ce qui fonctionne pour construire de l'aléatoire ?

Les écouter et leur laisser le choix est une nécessité de territoire. Les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent, disent-ils, conforter la commune comme cellule de base de la démocratie locale. Le citoyen doit être entendu. C'est par le maire et les élus municipaux qu'il l'est le mieux. C'est dans une politique municipale qu'il s'investit. Peu de citoyens connaissent les élus des autres institutions ou collectivités. Ne parlons pas des élus communautaires ou, pire, métropolitains. Comme le soulignait Bruno Retailleau, la confrontation dans les politiques locales est essentielle. Selon lui, « l'élu doit être à portée d'engueulade C'est pourquoi j'aurais souhaité que le champ d'application de cette proposition de loi soit plus large et touche l'ensemble des communes, qu'elles soient membres d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, quand le groupe écologiste inscrit à notre ordre du jour une proposition de loi dont l'objet est l'effectivité du droit à l'eau potable et à l'assainissement pour tous, il est accusé par la droite sénatoriale de manoeuvre électorale. égard au procès d'intention qui nous a été fait hier, que rétorquer aujourd'hui à cette même droite sénatoriale lorsqu'elle propose un texte d'affichage sur le thème de l'eau ? ? Il est évident que la présente proposition de loi envoie un message clair aux élus locaux, autrement dit aux grands électeurs, à l'approche du renouvellement partiel de notre assemblée, au mois de septembre En effet, avec cette proposition de loi, vous vous targuez, mes chers collègues, de revenir sur la réforme du bloc communal, en écartant le caractère obligatoire du transfert des compétences en matière d'eau et d'assainissement des communes aux communautés de communes dont elles sont membres.

En ce sens, l'exemple de la compétence « eau » est particulièrement édifiant. En effet, le régime juridique est issu d'un accord entre le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Olivier Dussopt, du groupe

Sur le fond, votre proposition de loi tend à écarter le caractère obligatoire, à compter du 1 janvier 2020, du transfert des compétences des communes en matière d'eau et d'assainissement aux communautés de communes dont elles sont membres. Nous comprenons que cette modification des compétences communales interpelle les élus locaux. Toutefois, n'oublions pas qu'il faut parfois forcer le destin pour obtenir des évolutions souhaitables de notre droit positif. En effet, rétablir la liberté, pour les communes, de transférer ou non certaines de leurs compétences ne nous paraît pas opportun. D'une part, cela induirait un manque de cohérence juridique d'un territoire à l'autre.

de cohérence juridique d'un territoire à l'autre. D'autre part, le niveau de l'intercommunalité nous paraît le plus adapté pour gérer les compétences « eau » et « assainissement », et ce à plusieurs égards. Tout d'abord, mutualiser la gestion de ces deux compétences au niveau des communautés de communes permet, par définition, de réaliser des économies d'échelle. Ces dernières sont bienvenues quand on sait les contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités locales- il en a longuement été

dernier. Dans le même ordre d'idées, il ne faut pas oublier que l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » coûte cher et peut constituer un véritable poids pour les petites communes. Ces dernières ne sont alors pas en mesure de gérer directement en régie ces services publics et sont souvent contraintes de les déléguer

Surtout, la conséquence de la délégation de service public, pour les collectivités, est double : premièrement, le recours au privé coûte cher aux communes et aux habitants, qui voient leurs factures augmenter ; deuxièmement, on dépossède les élus locaux de leur capacité de mise en oeuvre et de gestion d'un service public fondamental. Ainsi, la mutualisation à l'échelle intercommunale permettrait de pallier ces difficultés. Enfin, retenir le niveau de l'intercommunalité est également avantageux du point de vue de l'usager. le prix de l'eau varie d'une commune à une autre. La mutualisation à l'échelle intercommunale, en plus de diminuer les coûts de gestion, entraînera un rééquilibrage des tarifications, et donc des factures d'eau. Pour le groupe écologiste, le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes est le fruit d'un compromis politique auquel la droite sénatoriale

Sueur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il faut être clair : la loi NOTRe a été adoptée par la majorité du Sénat et de l'Assemblée nationale.

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, prévoit que les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement seront obligatoirement transférées des communes aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1 janvier 2020. Aujourd'hui, en droit positif, l'eau et l'eau et l'assainissement constituent pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération des compétences optionnelles, à la différence des communautés urbaines et des métropoles, pour lesquelles elles sont obligatoires. En pratique, la gestion de ces services publics est assurée par les communes dans plus de 73 % des cas concernant l'eau potable, 88 % concernant l'assainissement collectif et 53 % concernant l'assainissement non collectif. Cet état des lieux explique, pour partie, la très forte opposition des élus locaux à ces nouveaux transferts de compétences obligatoires. Ceux-ci craignent surtout, de façon fondée et justifiée, que ces

À l'heure actuelle, dans de nombreuses communes, les services relatifs à l'eau et à l'assainissement sont financièrement gérés avec une très grande frugalité. Dans nos communes rurales, ils sont assurés de façon bénévole ou quasi bénévole par des élus municipaux, ainsi que par des agents communaux polyvalents ou à temps non complet. Or la prise en charge systématisée de l'eau et de l'assainissement par les communautés de communes et les communautés d'agglomération impliquera nécessairement la mise en place de services intercommunaux, avec le recrutement de personnels et, par là même, l'engagement de nouvelles dépenses de fonctionnement importantes. Dans le même ordre d'idée, le contexte financier et budgétaire étant extrêmement contraint, conjugué à toutes les obligations anciennes ou récentes qu'elles doivent déjà assumer, les intercommunalités ne sont pas toutes en mesure d'assumer de façon satisfaisante la gestion des services de l'eau et de l'assainissement. Bien au contraire, ces nouveaux transferts de compétences à marche forcée- cette expression a été prononcée précédemment !- risqueraient de déstabiliser fortement une organisation territoriale qui est, dans l'ensemble, satisfaisante, mais également économe en fonctionnement.

de déterminer librement quel est le niveau territorial le plus pertinent ou le plus à même de mener au mieux une mission de service public, avec la plus grande efficience fonctionnelle ainsi que financière. C'est inscrit dans Aussi, pour toutes ces raisons, il ne semble pas pertinent de devoir imposer un seul et même modèle d'organisation dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, mais plutôt de faire confiance à l'intelligence des élus locaux, afin qu'ils s'organisent de la façon qui leur semblera la plus adaptée pour leur territoire. C'est pourquoi il est préférable que ces compétences

que nous avons votée, veuille corriger à la marge un certain nombre d'excès, ressentis comme tels sur le terrain. Pour terminer de façon plus générale sur l'intercommunalité, il est évidemment indispensable de mutualiser les énergies- je ne reviens pas sur cette évidence !- et d'optimiser les dépenses publiques de chaque territoire. Néanmoins, mes chers collègues, soyons vigilants à ce que tous les bienfaits apportés par les communes à notre pays, et qui lui donnent son « âme », ne disparaissent pas avec le développement d'une intercommunalité de plus en plus grande et intégrée, génératrice d'économies et d'efficacité, lesquelles restent d'ailleurs

n'oublions jamais que la proximité est une condition de la réussite de la vie en société et que c'est dans « la commune que réside la force des peuples libres » et que « si le pouvoir vient d'en haut,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comment vous convaincre en trois minutes de ne pas voter cette proposition de loi ? tient à la crédibilité de la loi et du législateur. Comment justifier la modification de la loi du 7 août 2015 à peine un an et demi après son adoption ? C'est une mauvaise besogne, après avoir déjà, à l'article 18-1 de la loi Montagne, vidé de sa substance le transfert de la compétence tourisme et après avoir tenté de faire de même voilà quelques mois, entre départements et régions, pour la compétence transports scolaires.

au moment de la montée en puissance des métropoles et des grandes régions. Ou alors trouvez une autre cohérence et proposez la suppression des métropoles et des grandes régions

de semer le doute et de dire qu'il faut tout arrêter parce que la loi pourrait changer ? Ce texte est, me semble-t-il, contre-productif ! La quatrième raison tient à l'intérêt des collectivités locales. Le fond de la présente proposition de loi laisse penser qu'il y a une concurrence entre les communes et les intercommunalités et que le caractère obligatoire des nouvelles compétences représenterait un risque pour l'échelon communal. Sous couvert du sauvetage du soldat communal, n'affaiblissez pas son meilleur rempart, l'intercommunalité ! L'élu intercommunal, vous le savez, mes chers collègues, est d'abord un élu communal. Le bloc local- la commune alliée à son intercommunalité -doit être renforcé pour trouver sa place dans le nouvel ordre régional et métropolitain. Tel est le véritable enjeu, que nos territoires soient urbains, périurbains ou ruraux. ma conclusion, madame la présidente. Accessoirement, mais ce serait un autre débat, je crois que les agences de l'eau seraient les premières à se réjouir du vote à venir,

que le Sénat se soit saisi de la présente question en cette fin de session, avec l'examen de la proposition de loi visant à maintenir les compétences « eau » et « assainissement dans les compétences optionnelles des communautés de communes, qui sera, je le souhaite, complétée par l'adoption de l'amendement de notre collègue Alain Joyandet tendant à élargir ce texte aux communautés d'agglomération ; j'y souscris totalement. Malgré un calendrier progressif, les compétences « eau » et « assainissement » seront attribuées obligatoirement aux communautés de communes et d'agglomération à compter du 1 janvier 2020. je trouve qu'il est intelligent d'amender une loi quand on se rend compte qu'elle ne correspond pas ou n'est pas adaptée aux besoins des communes. Je souhaite m'attarder sur la question prégnante de la gestion des eaux pluviales urbaines, qui n'a jamais été abordée dans les débats, sauf par vous, monsieur le ministre, dans votre propos Et pour cause, c'est une note de la Direction générale des collectivités locales du 13 juillet 2016 qui est venue préciser les contours des compétences dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, mentionnant que la compétence assainissement incluait la gestion des eaux pluviales. Le Conseil d'État, dans une décision du 4 décembre 2013, assimile la gestion des eaux pluviales à un service public relevant de la compétence « assainissement ». Ainsi, il n'y a pas de distinction selon le mode d'exercice de la compétence « assainissement », qu'elle s'exerce à titre optionnel ou obligatoire.

sujet fort complexe !-, il eût été pertinent de disposer d'un retour d'expérience avant d'ajouter obligatoirement l'assainissement et les eaux pluviales. Rappelons que le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » n'était pas prévu dans le texte initial. Il a été introduit par le Gouvernement, sans évaluation préalable des effets au niveau local ni concertation. Aucune étude d'impact n'a été réalisée pour déterminer les enjeux et les conséquences d'un tel transfert, pas plus que sur l'organisation, le fonctionnement, le prix de l'eau ou la gouvernance locale. Nous avions été nombreux sur ces travées à nous opposer à ce transfert imposé, augurant qu'il n'apporterait aucune amélioration en termes d'organisation, mais plutôt une désorganisation des structures, une inégalité territoriale, une gestion de l'eau et de l'assainissement hétérogène à l'intérieur d'un même périmètre. Plutôt que de faire confiance aux élus pour décider de l'organisation la mieux adaptée aux enjeux et contraintes qu'ils rencontrent dans leurs territoires, le Gouvernement a imposé une fois de plus un modèle unique. Si, sur certains territoires, le transfert des compétences peut s'avérer pertinent, cela ne peut être une généralité territoriale. Le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » fait fi des réalités et paramètres locaux, des infrastructures existantes, des moyens d'exploitation des services, des volontés politiques locales, et ne peut qu'entraîner des complexifications administratives, avec un impact sur les coûts, à la charge des usagers. Dans un contexte budgétaire contraint et avec la mise en place de nouveaux transferts de compétences, les collectivités ne pourront assumer ce transfert Je souhaite citer mon département en exemple. Depuis 1952, un syndicat regroupe 463 des 469 communes de Charente-Maritime, acteur majeur dans le domaine de l'eau, véritable service départemental de l'eau. Son fonctionnement a pour principe la mutualisation des ressources en eau interconnectées, des moyens techniques d'exploitation, des ouvrages de production et de distribution, et la péréquation du prix de l'eau à l'échelle départementale. En Charente-Maritime, le partage de l'eau entre usages domestiques, agricoles, ostréicoles et touristiques est très complexe. Cette gestion mutualisée permet une solidarité intégrale des territoires ruraux, urbains et littoraux. Dans sa rédaction actuelle, la loi NOTRe pourrait favoriser le retrait des EPCI urbains denses au détriment des zones rurales et désorganiser les conditions d'approvisionnement en eau, les services d'exploitation et les secours réciproques entre territoires. la multiplication inutile de points de vente d'eau en gros et une perte de réactivité en cas de crise climatique. Plus globalement, l'alimentation en eau potable doit être réfléchie à l'échelle des bassins versants hydrographiques pour les eaux de surface ou de bassins d'alimentation hydrogéologique pour les eaux souterraines. Il est rare que les périmètres naturels correspondent aux limites administratives des EPCI à fiscalité propre. Enfin, il conviendra d'être vigilant sur le respect du principe de représentation-substitution, qui permet de préserver les grands syndicats en cas de prise de compétence par un EPCI, même de façon optionnelle. Si nous ne revenons pas sur ce transfert « obligatoire », nous allons, au mieux, déstabiliser des organisations qui fonctionnent très bien et doivent être consolidées au regard de leur rôle indispensable en termes de solidarité Néo-Aquitain, je suis bien entendu plus girondin que jacobin. Je soutiens qu'il faut faire confiance aux élus de proximité et leur laisser la gestion des compétences qu'ils sont les plus à même de réaliser dans leurs territoires- nous en avons la preuve tous les jours. Je voterai donc en faveur du maintien de l'eau et de l'assainissement dans les compétences optionnelles des communautés de communes ou d'agglomération. Très bien ! La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Quatrièmement, en montagne, les compétences « eau » et « assainissement » répondent à des logiques de bassins, c'est-à-dire des logiques naturelles qui enferment les réseaux sans intérêt de maillage, et non dans des logiques administratives.

de la très grande diversité des territoires de notre pays. Au sud de l'Aisne, un très gros syndicat, l'Union des services d'eau du sud de l'Aisne, prélève de l'eau dans la Marne pour la distribuer à plus de 60 000 habitants, après l'avoir traitée bien sûr. Dans le centre du département, une initiative ambitieuse est portée par la communauté de communes du Val de l'Aisne. Mais partout sur le territoire, de petits syndicats ou des syndicats de moyenne dimension, avec un très fort engagement des élus et, souvent, une part de bénévolat considérable, répondent à la demande des habitants.

aux acteurs des territoires de jouer l'efficacité ? Je ne voudrais pas que le Sénat décourage ces femmes et ces hommes qui donnent de leur temps.

J'aime beaucoup M. Desessard, qui a le verbe haut, mais je l'invite à traverser le périphérique pour venir voir des intercommunalités en province.

des sénateurs que nous sommes tous consiste à ausculter les territoires et de revenir à une juste proportion. La loi NOTRe a été adoptée, mais, comme toutes les lois, elle a des aspérités qu'il faut polir pour construire cet édifice qu'est la République française.

et économique. L'eau potable est diverse et elle ne peut pas être enfermée dans un carcan uniformisé pour tout le pays, et encore moins dans un carcan idéologique.

Je vous remercie

je vois mal comment on peut mettre en place un dispositif différent pour, d'une part, les communautés d'agglomération et, d'autre part, les communautés urbaines et les métropoles. Bien

d'un compromis, qui ne satisfait personne. Cela explique que nous revenions sur ce texte par toute une série de propositions de loi- celle-ci n'est pas la première et ne sera certainement pas la dernière.

des collectivités territoriales, le CGCT, prévoient actuellement le principe de l'équilibre des services publics industriels et commerciaux que sont les services publics de l'eau et de l'assainissement,

Toutefois, d'une part, l'eau et l'assainissement relèvent des compétences obligatoires des métropoles et, d'autre part, si la métropole d'Aix-Marseille-Provence, en vertu des compétences qui lui sont spécifiques, peut déléguer ces matières au conseil de territoire, c'est à l'exception

Je crois que le trophée de la tératologie administrative revient incontestablement à la métropole Aix-Marseille-Provence. ! Si l'on peut arriver à la faire fonctionner, ce ne sera pas plus mal. Ensuite, c'est le problème qui se posera avec les fameuses communautés « XXL

et le groupe écologiste- une fois n'est pas coutume, même si cela fait deux fois en peu de temps. Merci de votre soutien. Je veux dire à Jean-Pierre Sueur que j'ai admiré son numéro d'équilibriste, mais je connais son talent ; cela ne m'a donc pas étonné de sa part.

dans un esprit constructif, dans la volonté républicaine de porter des textes qui soient bien ficelés et bons pour nos collectivités et nos concitoyens.

avec nous, parfois contre nous, mais toujours dans une vision commune de l'intérêt général et de l'intérêt de la France.

le Sénat va suspendre ses travaux en séance publique, en laissant le soin à notre président de le convoquer s'il y avait nécessité. Cette suspension ne concerne que nos travaux en séance publique. Durant cette période, notre assemblée poursuivra les divers travaux engagés au sein de ses commissions, délégations, missions d'information et commissions d'enquête. Le programme prévisionnel de ces travaux, qui vous a été communiqué le 13 février dernier, figure sur le site internet du Sénat. Personne ne